Cette aide universelle d'urgence vise à combler un réel manque lorsque les victimes de violences conjugales rencontrent des difficultés à s'extraire de l'emprise de leur conjoint violent en raison de leur dépendance financière,

résultat de nos nombreux échanges avec les associations compétentes, les travailleurs sociaux, les services de gendarmerie et de police, le procureur et la caisse d'allocations familiales. Ce travail de terrain

qui a su s'emparer de ce texte, en comprendre les enjeux et l'enrichir utilement lors de son passage en commission. Le Président de la République a fait des droits des femmes et de la lutte contre les violences faites aux femmes l'une des grandes causes de son À ce titre, le 3 septembre 2019, le Gouvernement lançait le Grenelle des violences conjugales, qui déboucha sur un plan d'action global et inédit. Mme Élisabeth Borne, Première ministre, a renouvelé l'engagement du Gouvernement en faveur de cette cause. Il le faut, car les chiffres sont glaçants ! En 2020, en France, hors homicides, les forces de sécurité ont enregistré 159 400 victimes de violences conjugales commises par leur partenaire, soit une hausse de 10 % en un an. En 2021, quelque 143 morts violentes au sein du couple ont été recensées, contre 125 l'année précédente, soit 18 victimes en plus. Dans l'arrondissement de Valenciennes, le territoire dans lequel nous avons imaginé cette aide, les statistiques du parquet sont particulièrement inquiétantes. Chaque année, le service d'aide aux victimes accompagne 1 000 victimes de violences conjugales. En 2021, les services de police et de gendarmerie ont eu à traiter en moyenne 8 cas de violences intrafamiliales chaque jour. Face à ce constat alarmant, il est plus que nécessaire de s'interroger sur la façon de prévenir ces violences, d'anticiper, de protéger et d'agir en amont.

Il est également urgent d'apporter une réponse adaptée et rapide à ces victimes une fois l'emprise du conjoint violent malheureusement établie. Aider une victime qui trouve la force d'aller porter plainte, de demander une ordonnance de protection et de quitter le foyer conjugal-

très peu de temps après l'avoir quitté, faute d'autonomie financière immédiate. Ce constat, mes chers collègues, est celui des professionnels de terrain. J'ai souhaité faire de ce dispositif une aide universelle, le prêt octroyé n'étant pas soumis à des conditions de ressources ou à un statut particulier.

L'objectif est donc de garantir aux victimes les conditions financières nécessaires pour leur permettre de se libérer le plus vite possible de l'emprise. C'est pourquoi le dispositif répond également

S'inspirant des mécanismes extralégaux d'action sociale de la branche famille, le montant retenu pour cette avance d'urgence, versée en trois mensualités maximum, équivaut au revenu de solidarité active.

Si besoin était d'en justifier, son impact budgétaire sur les finances publiques est sans commune mesure avec les conséquences financières d'une mise à l'abri de la victime et de ses enfants. En effet, un

L'idée est simple : faire payer l'auteur des violences pour une situation dont il est responsable. Enfin- il s'agit là d'une condition essentielle d'efficacité du dispositif proposé le président du conseil départemental sera informé dès la transmission de la demande à la CAF, afin d'engager immédiatement l'accompagnement social de la victime, parallèlement au versement de l'aide Concrètement, cela signifie un accompagnement global de la victime, dès le dépôt de plainte, l'ordonnance de protection ou le signalement par un travailleur social. Ce dernier fera office de personne-ressource tout au long du parcours de rebond de la victime. En effet, rappelons-le, l'objectif est non seulement de sécuriser les situations fragiles, mais aussi, et surtout, de conduire à une indépendance pérenne. Cela passe forcément par un accompagnement multidimensionnel. Logement, démarches administratives, accompagnement juridique, accompagnement santé et psychologique, insertion professionnelle : autant de domaines dans lesquels les travailleurs sociaux des départements et des centres communaux

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, quelle que soit notre place dans l'hémicycle, quelles que soient nos convictions politiques, nous rejetons tous la violence. Ces violences conjugales détruisent la vie de trop nombreuses victimes et de trop nombreuses familles. Elles touchent toutes les catégories de notre société. Notre pays s'est toujours grandi à protéger les plus fragiles et les victimes d'actes de violence. Cette aide universelle s'adresse à l'ensemble des victimes de violences conjugales, quels que soient leur sexe, leur origine, leur statut ou leur âge. Elle se veut un moyen de rendre aux leur dignité et de leur permettre de relever la tête et de s'extraire d'une situation personnelle qui n'apporte que souffrance et douleur. Elle sera, je l'espère, si vous l'adoptez,

collègues, Valérie Létard a rappelé le contexte douloureux dans lequel s'inscrit cette proposition de loi. En dépit de la mobilisation des pouvoirs publics, les violences commises au sein du couple perdurent à un niveau élevé. Dans l'Hexagone, une enquête statistique estime à 295 000 le nombre annuel de victimes de violences conjugales entre 2011 et 2018, dont 72 % de femmes.

La proposition de loi entend répondre à cet enjeu et puise sa force dans les retours concrets d'expérience. Valérie Létard a en effet présenté le travail qu'elle mène avec le département et la caisse d'allocations familiales du Nord pour mettre en place un prêt d'urgence et un accompagnement global des victimes de violences conjugales identifiées par les services sociaux. Le texte est issu du constat empirique d'un déficit à combler dans les politiques publiques que nous déployons en faveur des victimes de violences conjugales. Il convient de les aider à quitter définitivement leur partenaire violent, en leur apportant une aide cruciale dans des délais très réduits. Les données issues des appels au numéro 3919 « Violences Femmes Info » montrent que 59 % des victimes souhaitent quitter le domicile conjugal, tandis que 18 % d'entre elles indiquent avoir effectué plusieurs départs du domicile. Il est donc très difficile pour la femme de réussir à couper définitivement les ponts avec son tortionnaire. La précarité économique ou les incertitudes financières figurent souvent parmi les freins au départ des victimes. Ces dernières peuvent être sans emploi ou sans prestations sociales, mais aussi disposer de ressources propres et en être privées par l'emprise économique dont le conjoint violent fait preuve. Les moyens employés par les auteurs de violences pour placer leur victime dans une dépendance économique sont nombreux : chantage financier, confiscation des ressources ou des moyens de paiement, comportements visant à placer la victime dans des surendettements personnels Dès lors, comment donner les moyens financiers aux victimes de s'extirper de leur environnement violent ? La proposition de loi choisit d'accorder une aide d'urgence, débloquée en trois jours et versée par la caisse d'allocations familiales pendant trois mois. Le besoin de créer une aide d'urgence est un constat partagé sur les travées de notre assemblée. Une proposition de loi à l'objectif similaire, déposée par notre collègue Michelle Gréaume, adaptait le régime existant du revenu de solidarité active pour permettre aux CAF de verser des avances sur droits supposés au RSA, financées par le département. La proposition de loi que nous examinons prévoit un dispositif, sous la forme d'un prêt qui se rapprocherait des prêts d'honneur que les conseils d'administration des CAF peuvent librement consentir au titre de leur politique d'action sociale.

Ce prêt à taux zéro serait versé en trois mensualités, dont la première devra être payée dans un délai très court- la commission l'a porté à trois jours ouvrés. Ce délai reste très ambitieux, mais l'étendre davantage aurait affaibli l'intérêt du dispositif d'urgence. du dispositif d'urgence. Le montant du prêt sera fixé par décret. Il reviendra au pouvoir réglementaire de prévoir des montants majorés lorsque la victime quitte le domicile avec ses enfants. J'insiste sur ce point, en présence de Mme la ministre : les enfants sont directement victimes des violences conjugales, et les femmes victimes quittent rarement le domicile en abandonnant leurs enfants. L'aide d'urgence devra donc être adaptée à la situation familiale des victimes. La commission s'est penchée sur la question des conditions d'octroi permettant aux victimes de violences conjugales de faire valoir leur droit. Elle a considéré qu'un fait générateur trop souple risquerait de gêner la mise en oeuvre de la loi et a donc retenu des conditions d'octroi précises. Elle a ainsi conditionné la délivrance de l'avance à une ordonnance de protection ou à un dépôt de plainte attestant de violences conjugales. Ces deux critères étaient déjà prévus à titre illustratif par le texte initial. Cependant, nous savons bien que nombre de femmes n'osent pas pousser la porte de la gendarmerie ou de la police et dénoncer les faits qu'elles subissent. De même, seules 5 800 ordonnances de protection ont été délivrées en 2021 par les juges aux affaires familiales. C'est pourquoi, afin de ne pas trop restreindre l'accès à ce prêt d'urgence, la commission a ouvert la prestation aux victimes de violences attestées par un signalement adressé au procureur de la République. S'appuyant sur une nouvelle disposition prévue par la loi du 30 juillet 2020 visant à protéger les victimes de violences conjugales, certains centres hospitaliers ont contractualisé avec le parquet, afin de faciliter, avec l'accord de la personne, les signalements des victimes prises en charge médicalement. L'avance d'urgence pourra ainsi s'appliquer à cette situation. L'article 1 prévoit également que les allocataires de l'avance bénéficient des droits accessoires à la prestation du RSA. À côté du dispositif financier, la victime doit pouvoir être aidée, comme c'est déjà souvent le cas, par les associations ou les travailleurs sociaux des collectivités locales. La commission a précisé que ces droits accessoires comprennent également un accompagnement social et professionnel adapté à leur situation, à l'instar de celui qui aux bénéficiaires du RSA. La commission a également adopté un amendement, déposé par notre collègue Victoire Jasmin, visant à permettre aux bénéficiaires de l'avance d'urgence d'être domiciliés de droit auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale ou d'un autre organisme agréé. Enfin, la commission a précisé les règles de récupération des avances, lesquelles seraient très proches des modalités déjà existantes pour les prêts consentis par les CAF. La dette pourra ainsi être remboursée en une ou plusieurs échéances si le bénéficiaire le souhaite. Sinon, elle sera récupérée par retenues sur les prestations sociales par ailleurs versées par les caisses. Ces dernières pourront décider de remises ou de réductions de créances. Cette possibilité n'est pas hypothétique : les conseils d'administration des caisses devront faire preuve de discernement pour ne pas ajouter une dette à des situations de précarité ou de surendettement. La proposition de loi prévoit également un mécanisme inédit de subrogation des CAF dans les droits des victimes de se constituer partie civile pour demander, en leur nom, la réparation du préjudice subi. Ce mécanisme ne serait applicable que lorsque les victimes renoncent à leurs droits, ce qui n'est pas une situation rare. La récupération de la créance de la CAF pourra alors se faire sur les dommages et intérêts prononcés au bénéfice de la victime, ce qui permettra de faire payer l'auteur des violences en lieu et place de la victime. L'article 2 de la proposition de loi prévoit des mesures ambitieuses, en disposant que la victime déposant plainte pour des faits de violences conjugales devra être informée par l'officier ou l'agent de police judiciaire de la possibilité de demander l'avance d'urgence. Plus encore, le gendarme ou policier « plaintier » devra enregistrer la demande de la victime et la transmettre à la CAF compétente, ainsi qu'au conseil départemental, chef de file de l'action sociale. Lorsqu'un travailleur social sera présent, cette mission lui sera naturellement assignée. Néanmoins, si le déploiement des intervenants sociaux en commissariat et unité de gendarmerie suit son cours, il est encore loin d'être effectif dans tous les départements. Nous nous sommes donc interrogés en commission sur le bien-fondé de cette disposition. À l'évidence, il ne s'agit pas là de compétences naturelles aux policiers et gendarmes. Nous avons cependant préservé cette possibilité de demander l'avance à l'occasion du dépôt de plainte. Nous savons tous Nous savons tous qu'une simple information des victimes sur leurs droits ne sera pas suffisante. Les personnes, souvent dans des états traumatiques, ne seront pas si nombreuses à aller d'elles-mêmes vers la CAF. En outre, les situations contraintes dans lesquelles elles se trouvent peuvent les empêcher de se rendre comme elles le souhaitent auprès d'un nouveau guichet, retardant alors le déclenchement de l'aide.

En outre, un amendement de coordination de la commission aura pour objet de permettre aux assistants d'enquête, que le projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur entend créer, d'exercer ces missions d'enregistrement et de transmission de la demande d'aide d'urgence. Voilà, mes chers collègues, le dispositif que le présent texte entend établir. Le Gouvernement a par ailleurs annoncé diverses mesures, notamment un « pack nouveau départ ». D'autres initiatives locales fleurissent : je pense à celle menée par la CAF du Var et le barreau de Toulon pour orienter efficacement les victimes de violences conjugales et mener sous quarante-huit heures un examen complet de leurs droits à prestations légales. Nous ne pouvons que nous réjouir que toutes ces avancées aillent dans la même direction. Le dispositif de cette proposition de loi n'est donc ni concurrent ni redondant. Il s'agit d'une occasion de compléter les dispositifs existants d'aide aux victimes de violences conjugales. C'est pourquoi la commission a adopté la proposition de loi. Il est évident que l'expérimentation dans le Nord pourra, le cas échéant, apporter des voies d'amélioration du texte en cours de navette parlementaire. Par ailleurs, elle lèvera sans aucun doute les réserves institutionnelles qui peuvent encore être formulées. Cette aide monétaire légale s'inscrira dans les environnements déjà formés par les acteurs de l'action sociale. Le texte laisse en effet la liberté au pouvoir réglementaire et aux parties prenantes de s'organiser au plus proche des besoins de chaque département. La parole est

La lutte contre les violences conjugales, premier pilier de la grande cause du quinquennat, s'est traduite par plusieurs actions concrètes, fruits pour la plupart du Grenelle des violences conjugales et du travail conjoint du Gouvernement et des parlementaires. C'est l'illustration que nous avançons collectivement sur ce sujet qui dépasse largement les clivages partisans. C'est aussi le résultat du ressaisissement collectif qu'a opéré notre société ces dernières années, notamment grâce à la vague #MeToo, qui a déferlé sur le monde. Nous ne pouvons que nous en réjouir. Trop longtemps, notre société n'a pas écouté les victimes, ne les a pas crues, les laissant souvent seules face à l'emprise, abandonnées face aux coups, dans un huis clos avec leur agresseur. Depuis cinq ans, nous n'avons eu de cesse de renforcer les dispositifs de protection ou d'en créer de nouveaux. Je pense aux téléphones grave danger, aux ordonnances de protection, aux aux bracelets anti-rapprochement, à la présence renforcée des intervenants sociaux dans les commissariats et les gendarmeries, à la formation massive des policiers, des gendarmes et des magistrats, mais aussi à la considérable nombre de places d'hébergement d'urgence durant le précédent quinquennat. Ce mouvement, je compte bien entendu le poursuivre. La Première ministre a annoncé le 2 septembre dernier qu'elle présiderait dans les prochains mois

Oui, je partage votre constat : il faut aider les femmes et les victimes à sortir de cette emprise.

Quant à votre texte, il vise à créer un dispositif d'aide financière sous la forme d'une avance versée par les caisses d'allocations familiales aux femmes victimes de violences. Il s'agirait d'un prêt sans intérêt,

à sécuriser les femmes pour qu'elles se décident à fuir. Pour répondre à cet enjeu, votre texte permet notamment à la CAF, un mécanisme de subrogation, de se retourner contre l'auteur des violences pour obtenir le remboursement du prêt. du prêt. Un tel dispositif se heurte néanmoins en droit au principe de la subrogation légale, qui suppose que les créances transmises soient de même nature et répondent au même régime juridique. l'avance octroyée par la CAF est un prêt sans intérêt, de nature et de régime distincts des indemnités octroyées par le tribunal correctionnel en réparation du préjudice subi par la victime de violences. La mise en oeuvre de ce dispositif serait donc d'une particulière complexité, et le remboursement par l'auteur semble très hypothétique. De manière plus générale, si l'autonomie financière est un volet essentiel de l'aide que nous devons apporter à ces femmes, il n'est pas le seul. Comme vous le savez, leurs besoins sont multiples logement, aide financière, accès aux droits, garde d'enfants, réinsertion professionnelle, accompagnement psychologique ... L'esprit du « pack nouveau départ » passe justement

Nous souhaitons y associer pleinement les parlementaires et nous inspirer des dispositifs qui fonctionnent sur leur territoire. J'aimerais d'ailleurs, comme vous l'avez fait, madame

Var a signé un protocole avec le barreau de Toulon pour prendre en charge sous quarante-huit heures toute victime de violences conjugales à la demande de son avocat, une aide financière étant versée aux victimes pour un relogement en urgence. La CAF du Val-d'Oise apporte des aides pour acquérir des biens d'équipement ménager ou mobilier de première nécessité. Dernier exemple, la CAF de la Somme finance une aide au départ d'urgence d'un montant de 500 euros, plus 200 euros par enfant, versée aux femmes victimes de violences conjugales par les associations têtes de réseau départemental.

et qui a inspiré votre proposition de loi, est intéressante. Elle peut être intégrée dans les réflexions du Gouvernement, mais elle doit être, à notre avis, enrichie pour couvrir tous les besoins des femmes.

C'est le cas des violences conjugales, parce qu'il s'agit de situations où la violence s'immisce dans l'intime, où l'amour s'abîme dans l'horreur et dans la haine, où les problématiques sont aussi complexes que révoltantes. Cette précaution ne doit pas nous empêcher d'agir, bien au contraire. Seulement, il convient de privilégier la voie du pragmatisme à celle de l'idéologie, la mesure et l'action aux condamnations à l'emporte-pièce. C'est pourquoi je tiens à saluer l'initiative de notre collègue Valérie Létard, dont le travail répond précisément à cette exigence. Que le dispositif de la proposition de loi soit directement inspiré par une expérimentation conduite par des acteurs de terrain a de quoi nous rassurer à cet égard. Ces acteurs de terrain, qu'il s'agisse des services sociaux de proximité ou des associations de soutien aux victimes de violences conjugales, sont unanimes sur la question : le soutien aux victimes doit passer par une aide d'urgence, facilement accessible et rapidement décaissable. En effet, comme je le disais en préambule, les victimes de violences conjugales sont particulièrement fragiles et précaires, puisqu'elles partagent bien souvent le même domicile et les mêmes revenus que leur bourreau. En conséquence, les victimes n'ont aucun moyen d'échapper à ces violences, qui sévissent au sein même du foyer. D'où le cercle vicieux de la violence, qui s'installe de manière pernicieuse dans la normalité d'un couple, où les sévices, tout d'abord isolés, commencent à se répéter, puis à devenir de plus en plus graves. Et puisque les victimes n'ont pas les moyens de s'échapper, ces violences finissent par se banaliser : elles deviennent régulières, bien souvent quotidiennes ; bientôt, les victimes ne peuvent plus s'y opposer ni même les éviter. Que faire face à cette banalisation du mal ? Que faire, alors même que les victimes ont parfois tendance à occulter ou à nier les violences qu'elles subissent, parce qu'un lien affectif les unit encore à leur bourreau ? La proposition de loi que nous allons examiner vise précisément à offrir à ces victimes l'espoir d'une échappatoire. En prévoyant la possibilité de débloquer en trois jours un pécule pour permettre à la victime de se mettre à l'abri, nous apportons une réponse concrète pour briser ce cercle vicieux de la violence. En commission, j'ai fait part de plusieurs interrogations relatives à la sécurisation du dispositif, notamment pour ce qui concerne les modalités de versement de l'avance et de son recouvrement. Je crois que l'adoption des amendements proposés par la rapporteure a contribué à renforcer le dispositif. Les précisions apportées, notamment pour mieux définir les critères d'octroi, rendront le dispositif envisagé plus efficace et plus opérant. Pour dire clairement les choses, c'est toute la difficulté de ce dispositif qui doit apporter une réponse rapide pour faire face à l'urgence d'une situation, en évitant à tout prix que l'irréparable ne se produise. C'est cet objectif qui nous oblige à veiller, en priorité, à la célérité du dispositif. Cela n'exclut pas une forme de contrôle, mais il est nécessaire que ce contrôle intervienne, c'est-à-dire après le versement de l'avance, afin de ne pas ralentir une procédure dans laquelle la mise à l'abri d'une victime tient parfois à peu de chose. je crois que le travail en commission a amélioré une initiative parlementaire de grande qualité, qui répond aux préoccupations issues du terrain. Nous avons déposé un amendement qui vise à répondre à un angle mort de la proposition de loi et qui a pour objet le versement par les mutuelles sociales

Depuis lors, des lois ont été votées en 2014, 2018 et 2020 pour tâcher de pallier nos manquements. Mais la France continue d'être un pays où les femmes meurent et sont victimes de violences, parce qu'elles sont des femmes. Le décompte de nos mortes est à 102 féminicides pour 2022. Nous ne cessons de dire tous les ans en novembre et en mars à toutes les victimes de violences que nous les croyons. Croire la parole est essentiel, mais, quand on est cru, encore faut-il pouvoir partir de chez soi, fuir son conjoint violent, en avoir la possibilité économique. Nous vivons encore dans un monde où la réalité est que, dans les couples hétérosexuels, la majorité des hommes gagnent plus d'argent que leurs conjointes, l'écart de revenus étant de 47 % en faveur des hommes. Cet écart se creuse avec les séparations conjugales.

femmes devront, sauf exception, rembourser ce prêt. Enfin, même si la procédure aboutit à une condamnation, la CAF pourra utiliser les dommages et intérêts obtenus pour réparation de violences,

Cela dit, le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires votera en faveur de ce texte, qui constitue malgré tout une avancée, un petit

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, 213 000, c'est le nombre de femmes qui déclarent avoir été victimes de violences physiques ou sexuelles par leur conjoint ou ex-conjoint sur une année. Les chiffres, nous le savons, sont plus qu'alarmants.

Elles sont toujours, lorsque l'issue n'est pas mortelle, source d'isolement et de vulnérabilité chez la victime, trop souvent livrée à elle-même, seule face à son bourreau. Face au calvaire que vivent de trop nombreuses victimes, nous devons agir. Agir, en protégeant les personnes victimes de violences conjugales. C'est l'ambition de la loi de 2010 que le Parlement et le Gouvernement ont renforcée sous la précédente législature et qui permet au juge des affaires familiales de statuer sur des mesures de protection sans que la personne ait déposé plainte. Le nombre d'ordonnances n'a cessé d'augmenter depuis 2015 ; il a même doublé en cinq ans. Agir, en éloignant le conjoint violent, car ce ne doit pas être systématiquement à la victime de quitter le domicile. C'est l'objectif du bracelet anti-rapprochement, dispositif de surveillance électronique créé par la loi du 28 décembre 2019, qui permet de géolocaliser la victime et son agresseur, ce qui constitue l'une des mesures les plus protectrices en matière de violences conjugales. Je pense également à l'instauration du référé violences conjugales, procédure qui permet au juge d'ordonner l'éviction du conjoint violent et l'attribution du domicile conjugal à la victime. Agir, en apportant assistance aux victimes en situation de vulnérabilité et en grave danger. C'est la raison pour laquelle le dispositif téléphone grave danger, accessible sept jours sur sept, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, a été généralisé, afin de permettre à toutes les victimes de violences conjugales d'y avoir accès sur l'ensemble du territoire. Il permet d'alerter et de faire intervenir immédiatement, grâce à la géolocalisation, les forces de l'ordre en cas de menaces ou de violences. Un numéro unique, le 3919, a par ailleurs été déployé, et l'examen de cette proposition de loi doit nous permettre d'en faire la promotion à destination de toutes les femmes victimes ou en danger. Agir, enfin, pour l'avenir des victimes. C'est tout l'objet du pacte Nouveau départ, annoncé en septembre dernier par Mme la ministre, qui accompagnera les victimes de violences de façon globale grâce à la mobilisation d'aides sociales, l'accès à la formation, l'aide au retour à l'emploi, l'hébergement d'urgence ou encore un soutien psychologique. Pourtant, malgré ces avancées salutaires et l'action du Gouvernement, la situation est critique, mes chers collègues. Trop de femmes, par peur de se retrouver seules avec leur conjoint violent, s'enferment dans le déni, parfois la honte, et renoncent à porter plainte ou à s'enfuir.

Le groupe RDPI partage son objectif, puisque le dispositif permettra à la victime de s'extraire, avec ses enfants, d'une situation de danger, en lui apportant une aide garantissant son autonomie financière. Protéger la mère, c'est aussi protéger les enfants. Ces enfants sont en effet les victimes directes, lorsqu'ils sont eux-mêmes frappés ou menacés, ou indirectes, lorsqu'ils sont tout simplement exposés à ces violences. Par ailleurs, ils sont souvent instrumentalisés pour maintenir une certaine emprise du conjoint violent sur la victime. Les études récentes montrent que les enfants traumatisés par ces violences ont davantage de problèmes de santé, comme des retards de croissance, et qu'ils présentent dix à dix-sept fois plus de troubles du comportement que les enfants qui vivent dans un foyer sans violence.

Mais je ne doute pas que Valérie Létard nous apportera des réponses complémentaires visant à pallier les difficultés que ce dispositif pourrait entraîner. En tout état de cause, et malgré cette réserve, notre groupe soutiendra sans réserve cette proposition de loi.

Celles et ceux d'entre nous qui ont déjà eu l'occasion d'accompagner des victimes de violences conjugales le savent : l'un des premiers écueils à la dénonciation des violences subies est la crainte des conséquences de cette dénonciation, en particulier le fait de devoir quitter le domicile

les restrictions aux modalités d'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite et d'hébergement de l'auteur des violences ; l'exclusion de la résidence principale de l'enfant chez l'auteur des violences ; l'augmentation de la durée et de la portée de l'ordonnance de protection ; la dissimulation de l'adresse protection ; la dissimulation de l'adresse de résidence et de l'école des enfants à l'ex-conjoint violent ; le renforcement de la lutte contre les violences post-séparation, etc. Je ne

sur les 9,06 milliards d'euros du budget total de la justice, [ ...] de 8,6 milliards d'euros sur les 13,1 milliards d'euros du budget total des forces de l'ordre, de 2,3 milliards d'euros sur les 16,1 milliards d'euros du budget total des urgences et des hospitalisations qui s'ensuivent. À cela, il faut ajouter le coût humain et social de ces infractions à la loi, puisqu'il y a, derrière ces actes, des vies brisées ». Plus de 200 000 femmes sont victimes chaque année de violences de la part de leur conjoint ou ex-conjoint. Sur la totalité des violences conjugales, 96 % des auteurs sont des hommes. Cela représente, pour nos finances publiques, un coût de 3,3 milliards d'euros par an. Au regard de ce que nous coûte la violence masculine, le budget que nous propose de mobiliser Valérie Létard est bien minuscule,

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le sujet des violences conjugales revient régulièrement devant notre assemblée, et force est de constater qu'il reste beaucoup à faire pour éradiquer ce mal qui ronge notre société. Le Nord est le deuxième département de France métropolitaine le plus touché ; c'est dire si Valérie Létard et moi connaissons bien la problématique. Une réalité locale qui rejoint les statistiques nationales des violences faites aux femmes. En 2019, selon l'Observatoire national des violences faites aux femmes, 213 000 femmes ont été victimes de violences physiques et sexuelles commises par leur partenaire ou ex-partenaire. Selon le bilan du ministère de l'intérieur paru cet été, le nombre de féminicides a augmenté de 20 % en 2021 par rapport à l'année précédente 122 de nos soeurs, de nos mères, de nos cousines, de nos voisines, de nos filles sont décédées sous les coups d'un conjoint ou ex-conjoint, contre 102 en 2020. Ce qui retient les femmes de quitter le domicile conjugal, outre l'emprise exercée par le conjoint, c'est le manque de ressources financières. En effet, il est fréquent que les victimes n'aient pas accès au compte bancaire du foyer ou qu'elles n'aient pas de source de revenus personnelle. Le départ est alors synonyme de difficultés à assurer, pour elles et pour leurs enfants, les achats de première nécessité. Très souvent, ces difficultés contribuent à un retour contraint au domicile conjugal. La mise en place d'une aide financière d'urgence aux victimes permettra d'encourager cette démarche salvatrice J'avais moi-même formulé cette proposition dans un texte déposé en février 2021 : il s'agissait d'attribuer le RSA en urgence aux victimes de violences intrafamiliales. Ce dispositif sera d'ailleurs expérimenté dès le mois prochain dans mon arrondissement du Valenciennois, sur l'initiative du département du Nord. On pourra au passage regretter que l'évaluation de cette expérimentation n'ait pas été attendue avant de débattre d'un dispositif alternatif. Dans le texte qui nous est soumis, l'aide prend la forme d'un prêt accordé par les caisses d'allocations familiales, déclenché dans un délai porté à trois jours ouvrés par la commission et versé en trois mensualités. Les modifications apportées par la commission ont permis de cadrer les conditions d'accès à cette aide sans qu'elles soient trop restrictives, et nous devons l'en remercier et saluer le travail de notre collègue Guidez, en tant que rapporteure de ce texte. Ce principe de soutien au départ d'urgence n'a pas vocation à remettre en cause le principe d'éloignement des auteurs des violences ni à résoudre à lui seul l'ensemble de la problématique des violences faites aux femmes. Je rappelle que les associations féministes demandent un investissement massif, à hauteur d'un milliard d'euros, afin d'engager efficacement une véritable lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants dans l'esprit de la grande cause nationale décrétée et annoncée par le Président de la République à l'aube de son précédent mandat. La prévention et la protection des femmes et des enfants victimes de violences sont également indispensables pour éviter que ces comportements ne se reproduisent de génération en génération. Néanmoins, il s'agit d'un premier pas, qui doit être salué, pour accompagner les victimes de violences conjugales. Avec cette proposition de loi, le Sénat a l'occasion d'envoyer un signal, en montrant que nous sommes capables de nous réunir et de dépasser nos divergences partisanes pour lutter contre les violences conjugales.

cinq ans que #MeeToo a libéré la parole des femmes, cinq ans que, avec courage, elles sont enfin sorties du silence, bravant le sentiment de honte qui trop souvent les enferme dans un carcan de culpabilité. Les témoignages se sont multipliés dans toutes les couches de la société, révélant au grand jour des violences jusque-là insoupçonnées ou ignorées. Les victimes se sont mises à parler et la société à les écouter- enfin Nous avons pris conscience de ce fléau. C'est une véritable révolution. Les violences conjugales sont un phénomène multiforme, complexe, qu'il nous revient de traiter dans sa globalité. Elles peuvent être physiques, psychologiques, mais aussi économiques. se traduisent dans les faits par une précarité telle que la victime ne peut survivre sans son agresseur. Chantage financier, confiscation des ressources financières ou des moyens de paiement, ces comportements visent à acculer la victime et à la pousser vers un surendettement personnel.

alors qu'une enquête statistique du ministère estime à 295 000 le nombre annuel de victimes de violences conjugales, dont 72 % de femmes et 28 % d'hommes- il ne faut pas oublier En 2021, quelque 122 femmes ont été tuées par un conjoint ou un ancien conjoint, soit une hausse de 20 % par rapport à 2020. J'ajoute qu'une étude de l'Institut national d'études démographiques de 2018 révèle que près d'une femme sur cinq se déclare en situation de violences conjugales en Martinique et en Guadeloupe. Un certain nombre de mesures ont déjà été prises ou renforcées : le téléphone grave danger- il y en a plus de 4 000 - ; le 3919 joignable sans interruption depuis le 30 août 2021 ; la messagerie instantanée qui permet de dialoguer avec un agent de police les plus de 9 000 places d'hébergement avec les 1 000 nouvelles décidées en début d'année ; les ordonnances de protection prises par un juge aux affaires familiales qui prononce l'éloignement du conjoint violent et permet, dans le même temps, d'organiser la vie de la famille les bracelets anti-rapprochement ; enfin, les centres de prise en charge des auteurs de violences pour éviter des récidives. Malgré ces avancées, les données issues des appels au numéro 3919 Violence Femmes Info montrent que 59 % des victimes souhaitent quitter le domicile conjugal et que 18 % d'entre elles indiquent avoir effectué plusieurs départs pour revenir au foyer faute de moyens financiers leur permettant d'être autonomes. Il leur est donc très difficile de couper définitivement les ponts avec leur tortionnaire, d'autant plus lorsqu'elles partent avec leurs enfants. L'aide financière d'urgence doit donc s'imposer comme l'un des piliers de la prise en charge et de l'accompagnement des victimes de violences conjugales. C'est une mesure de bon sens, qui émane du terrain, de celles et ceux qui travaillent au quotidien avec ces victimes

Quelques éléments du texte me semblent particulièrement importants. Nous savons que, au-delà de soixante-douze heures, les victimes, livrées à elles-mêmes, sont contraintes de rentrer au domicile. Ce dispositif répond à ce problème en versant, dans un délai maximum de trois jours, une somme dont le montant sera fixé par décret. Cette aide étant non pas une allocation, mais bien un prêt à taux zéro, elle devra être remboursée dans son intégralité selon un échéancier variable. Cependant, la proposition de loi contient un mécanisme permettant à la CAF de se constituer partie civile. Cela lui permettra, si le prêt est encore en cours moment du jugement, de se rembourser sur les dommages et intérêts versés par le coupable. Enfin, cette aide est universelle, et je pense que, à ce niveau d'urgence, il n'y a pas lieu de faire une quelconque distinction entre milieux sociaux. Nous connaissons tous le taux de non-recours aux aides sociales. C'est pour cette raison qu'il incombera soit à l'officier ou l'agent de police judiciaire, soit à l'intervenant social en commissariat et gendarmerie recevant la victime de l'informer de l'existence de ce prêt, d'en enregistrer la demande et de la transmettre à la CAF, ainsi qu'au conseil départemental, chef de file de l'action sociale. nécessitera une parfaite information et formation de ceux qui sont souvent en première ligne pour accueillir les victimes. Je terminerai mon propos en soulignant le travail formidable accompli par tous les partenaires, dans toutes les associations d'aide aux victimes de violences conjugales, souvent confrontées à des difficultés financières. Je garde en mémoire la lueur d'espoir qui se rallume dans les yeux de celles qui sont prises en charge et accompagnées pour se reconstruire et qui voient enfin leur avenir s'éclaircir. Je voudrais remercier chaleureusement notre collègue Valérie Létard d'avoir travaillé sur le terrain dans son département du Nord et concrétisé ce dispositif si utile, ainsi que Jocelyne Guidez de son travail consciencieux et sérieux de rapporteure, qui a permis d'amender ce texte avec précision. Je suis persuadée que cette proposition de loi permettra de réaliser un bond en avant dans la lutte contre les violences conjugales et pourra éviter bien des drames en offrant une échappatoire aux victimes. Il faut conclure, ma chère collègue. Le groupe Union Centriste votera évidemment en faveur de ce texte.

comme le souligne le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, « l'autonomie financière est une condition pour reprendre sa vie en main ». J'ajoute : lorsqu'il s'agit des femmes victimes de violences conjugales. Reprendre sa vie en main est un long parcours. Il faut tout d'abord que ces femmes soient écoutées et que l'on prenne en considération ce qu'elles disent, les mots et les souffrances qui les accompagnent. Elles cherchent aussi une protection pour, enfin, envisager de se reconstruire. La mise en place de cette avance d'urgence pour les victimes de violences conjugales incite à emprunter cette voie, si difficile soit-elle. une pierre qui s'ajoute à la construction d'une culture de la protection, si défaillante actuellement. Pour plus de 350 000 interventions par les forces de l'ordre au domicile des familles, seuls 79 000 79 000 procès-verbaux de renseignement judiciaire et mains courantes ont été déposés en 2019. La faille réside dans cet écart. S'il y avait eu une prise en charge à temps, on aurait pu éviter quelques victimes. dernier, j'ai rencontré Aïcha dans les locaux du foyer Louise Labé, géré par l'association Halte aide aux femmes battues, un centre d'hébergement spécialisé. Voici son témoignage : « Mon mari me frappait. Il me disait " Maintenant que tu n'as plus ta famille, je fais ce que je veux de toi ". Alors un jour, je suis partie avec un bébé dans le ventre, un dans les bras, mes claquettes et rien d'autre. Pendant deux ans, je n'ai pu toucher aucune aide. aucune aide. » Conjointement à la colère des femmes dont les signalements ne sont pas toujours entendus, il est heureux, si l'on peut s'exprimer ainsi, que l'actualité fasse écho au sujet qui nous réunit aujourd'hui. En réalité, la relative libération de la parole des femmes oblige les institutions à agir dans le bon sens : c'est ce que Il est temps que les victimes de violences conjugales soient guidées dans leurs démarches administratives et judiciaires, leur seul courage ne suffisant pas. Leur situation précaire et leur vulnérabilité, entretenues par des mécanismes d'emprise physique, psychologique et financière, aboutissent en fin de compte à leur isolement. Si elle est votée, cette aide, même insuffisante, sera d'une grande utilité, aussi bien pour les victimes de violences conjugales que pour leurs enfants. Je voterai en faveur de ce texte. La parole

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, il est difficile de ne pas partager l'ambition de cette proposition de loi déposée par notre collègue Valérie Létard, qui a eu l'amabilité de nous inviter à la cosigner, ce que plusieurs d'entre nous ont fait au sein du groupe RDSE. 143 victimes de morts violentes au sein du couple en 2021, dont 122 femmes. L'année 2022 ne semble malheureusement pas marquer de recul, ce qui a sans doute poussé le Président de la République à déclarer grande cause nationale du quinquennat, pour la seconde fois, la lutte contre les violences faites aux femmes. Le sujet a d'ailleurs fait la une des médias récemment, prouvant une fois de plus qu'aucun milieu n'était épargné par la violence et que, parmi les hommes politiques, certains avaient encore un long chemin à parcourir sur cette question. Poussés par la société civile et de nombreuses activistes, les pouvoirs publics tentent, avec des moyens et des résultats encore insuffisants, de réduire la violence au sein des couples. Le Grenelle contre les violences conjugales de 2019 a accouché de 54 mesures, dont 46 sont aujourd'hui en vigueur. Des outils existent, comme le téléphone grave danger ou le bracelet anti-rapprochement. En les assortissant d'un budget à la hauteur et en les accompagnant de mesures telles qu'une formation adaptée des forces de l'ordre ou l'éducation à la vie affective et sexuelle dès le plus jeune âge, nous pouvons espérer que la situation s'améliore dans les années à venir. Dans l'immédiat, et afin de compléter l'arsenal aujourd'hui disponible, cette proposition de loi vise à répondre à une problématique récurrente pour les victimes de violences conjugales : la dépendance financière. Elles sont en effet nombreuses à demeurer ou à retourner au domicile conjugal faute de ressources suffisantes, notamment lorsqu'elles ont des enfants à charge, qu'elles refusent naturellement de laisser derrière elles. Les aides, telles que le RSA, lorsqu'elles y sont éligibles, sont assorties d'un délai souvent rédhibitoire. Il est donc proposé, ici, de donner les moyens financiers aux victimes de s'extirper d'un environnement violent, en leur accordant une aide d'urgence, sous forme de prêt à taux zéro, délivré par la CAF en trois mensualités, dont la première débloquée sous trois jours. Cette avance est subordonnée à une ordonnance de protection délivrée par le juge, un dépôt de plainte de la victime ou un signalement d'un professionnel de santé adressé au procureur.

La victime n'aurait plus alors à rembourser le prêt. La PPL prévoit, par ailleurs, que les allocataires de l'avance bénéficient automatiquement des droits accessoires à la prestation du RSA, comme la complémentaire santé solidaire ou les droits décidés par les collectivités, tels que le tarif réduit pour les transports en commun.

Cette expérience sera particulièrement utile à sa généralisation. Une telle généralisation est souhaitable, voire indispensable puisqu'elle aboutira à la création d'un droit supplémentaire sur la question hautement sensible de la dépendance financière. Les auteurs de violences, eux, ne manquent pas de ressources. Le chantage financier et la confiscation des moyens de paiement sont fréquents. Ils aggravent le climat de violence, restreignent le champ de liberté des victimes et les éloignent de la perspective d'une fuite pourtant vitale. Pour toutes ces raisons, le groupe du RDSE votera d'une seule voix pour cette proposition de loi. La parole

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, que répondre aux victimes de violences, dont certaines, hélas, ne peuvent même plus nous entendre ? En tout état de cause, tous les mots prononcés dans cet hémicycle aujourd'hui n'apaiseront en rien la douleur des coups répétés d'un conjoint violent. Espérons néanmoins que ce débat puisse faire évoluer la cause des femmes et des hommes victimes de violences conjugales, afin que la peur change de camp une bonne fois pour toutes, qu'un véritable cadre protecteur et rassurant pour les victimes soit enfin mis en place, qu'elles ne se sentent plus seules et abandonnées à leur sort et qu'elles gardent ce qu'elles ont de plus précieux : leur liberté et leur dignité. Alors, le ton doit être humble, et la volonté politique ambitieuse ! Réunis pour examiner ce texte défendu par notre collègue Valérie Létard, nous ne pouvons que la féliciter pour sa proposition, qui va dans le bon sens rendre aux victimes de violences conjugales une indépendance financière, condition pour qu'elles se libèrent enfin des chaînes de l'angoisse de la violence. Ce texte est le fruit d'un consensus transpartisan. C'est avec honneur que j'en défends donc la teneur et en réaffirme la qualité. Le Sénat s'est saisi depuis de nombreuses années de ce sujet et demeure une source inépuisable de propositions lorsqu'il s'agit d'introduire des mesures efficaces et protectrices envers les victimes de violences conjugales. Le récent rapport sur les zones blanches de l'égalité doit appeler toute l'attention du Gouvernement sur la particularité, notamment, des zones rurales, qui apparaissent malheureusement comme des terreaux intarissables de féminicides. Si des moyens supplémentaires sont engagés pour endiguer cet effroyable fléau, il nous revient de veiller avec beaucoup de vigilance qu'ils puissent bénéficier à toutes et tous de façon et cela en tout point de l'Hexagone et des outre-mer. L'égalité entre les êtres, ce plébiscite de tous les jours, passe aussi par une égalité entre les territoires. Nous devons collectivement revoir notre copie pour que personne ne soit laissé sur le bord de la route. jours de la Journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes, affirmons d'abord notre reconnaissante admiration à celles qui ont trouvé les ressources pour demander de l'aide, entamer un processus de reconstruction et témoigner. Osons clamer enfin, car il le faut, que le combat pour l'égalité est une lutte de tous les instants, une bataille permanente, et que le moindre relâchement nous est interdit. Alors que les Françaises et les Français décompteront les heures avant le passage en 2023, d'autres procéderont déjà au décompte des femmes lâchement assassinées sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint. Le 1 janvier dernier, Muriel, Lisa et Éléonore ouvraient ce bal funeste illustrant les dysfonctionnements dramatiques de notre système judiciaire. Nous devons enfin comprendre que la non-assistance à personne en danger ne peut plus durer. preuve, un rapport de l'inspection générale de la justice de 2019 sur les homicides conjugaux indique que, si 41 % des victimes avaient alerté les forces de sécurité, 82 % des mains courantes et procès-verbaux de renseignement judiciaire n'avaient donné lieu à aucune investigation, tandis que 80 % des plaintes avaient abouti à un classement sans suite. Avant d'envisager d'autres réformes, il est urgent, pour celles qui sont encore en vie, d'appliquer les lois existantes. La responsabilité individuelle ne doit pas se diluer dans la responsabilité collective. La parole politique, la loi et la justice ont le pouvoir de remettre ce monde à l'endroit, ce monde où la victime a trop longtemps été la coupable. Et il nous faut penser au futur et ne pas hypothéquer la liberté de nos filles et de nos fils en laissant se perpétrer la violence devant eux, parce que ne pas arrêter la violence, c'est en engager une reproduction mécanique à l'égard de la génération suivante. Comment ignorer qu'un enfant témoin présente quatre fois plus de chance de devenir auteur de violences conjugales et six fois plus de chance de devenir victime ? Les études démontrent qu'ils subissent des traumatismes comparables à ceux que les personnes confrontées à la guerre développent. Comment tolérer encore en 2022 une telle destruction de l'enfance ? Il y a urgence à agir sur les plans de la détection, de la prise en charge et de la protection des victimes de violences, tout en s'assurant de la mise hors d'état de nuire des personnes violentes. Il est urgent de protéger, soutenir et accompagner celles qui sont, chaque jour, humiliées, esseulées et violentées. remercie de contribuer, grâce à vos travaux et aux dispositions de cette proposition de loi, à un meilleur accompagnement des victimes. Au-delà de ces avancées incontestables, la protection des victimes face aux violences doit rester une priorité collective. Le travail ne s'achèvera jamais tant qu'il y aura des êtres atteints

ce véritable fléau que constituent les violences conjugales ? Cette question, nous l'évoquons régulièrement au sein de cet hémicycle, tant le sujet est majeur, complexe et revêt plusieurs réalités. Le constat est unanime seule une mobilisation collective de tous les acteurs de la société permettra d'y arriver. Je souhaite ce matin rappeler trois chiffres : les violences conjugales ont augmenté de 20 % en 2021. 87 % des victimes de violences sont des femmes, mais seulement 3 % des victimes de violences conjugales avaient porté plainte en 2020. En février dernier, nous débattions ici même des mesures issues du Grenelle des violences Nous mettions alors en évidence l'importance d'une réponse judiciaire rapide et efficace, mais également la question de la sensibilisation et de la formation des professionnels, ainsi que le sujet ô combien essentiel

Même si le principe premier doit être l'éviction de l'auteur des violences, il convient de rappeler que 59 % des victimes souhaitent quitter le domicile. Une réalité, qui ressort des témoignages des victimes, s'impose on ne part pas ! ». La dépendance économique de certaines femmes demeure actuellement l'un des freins pour quitter le domicile conjugal. Par ailleurs, les violences économiques, qui vont du contrôle financier jusqu'à la dépossession totale de moyens financiers, sont souvent invisibles et mal identifiées. Ce type de comportement, qui fait partie intégrante des violences conjugales, mériterait

de faciliter et de sécuriser au mieux leur parcours. Aussi, je salue aujourd'hui cette proposition de loi et le travail mené par notre collègue Valérie Létard. Instaurer une aide universelle d'urgence pour les victimes de violences conjugales, c'est tout simplement une réponse concrète, qui peut se mettre rapidement en place- une réponse à un besoin identifié. Cette aide financière viendra ainsi compléter des initiatives locales qui ont émergé pour permettre d'accompagner les victimes sur le plan matériel. Je cite, pour exemple, l'association d'aide aux victimes Viaduq 67 dans le Bas-Rhin, qui distribue des produits de première nécessité aux femmes ayant quitté leur domicile. Je tiens à saluer le principe même de cette aide d'urgence, qui prendra la forme d'un prêt financier sans intérêt versé par les caisses d'allocations familiales. Je suis pleinement en accord avec les modalités envisagées par le texte, que le travail parlementaire a permis d'enrichir. Le mécanisme de subrogation des CAF dans les droits des victimes, pour demander réparation du préjudice subi et faire payer l'auteur des violences, me paraît tout à fait pertinent,

pour que le dispositif puisse fonctionner. Comme le souligne également l'auteure du rapport, cette aide d'urgence devra être accompagnée du déploiement d'intervenants sociaux en commissariat et unité de gendarmerie. Nous convergeons ici vers un constat déjà établi au moment du Grenelle : nous avons besoin de moyens humains au plus près des territoires, notamment dans la ruralité,

inspirée par des initiatives locales. Il s'agit là, à mon sens, de la meilleure manière de légiférer utilement et de manière pragmatique. À ce titre, je souligne le travail mené quotidiennement sur le terrain par les acteurs locaux, associations, élus locaux, parquets, services de police et de gendarmerie. Notre message collectif est clair : inciter les femmes à porter plainte, les encourager à dénoncer l'inacceptable et leur permettre de quitter le domicile, étape souvent cruciale et délicate, notamment lorsqu'il y a des enfants. Pour toutes ces raisons, le groupe Les Républicains salue ce texte et votera bien évidemment en sa faveur.

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, l'article 1 pose les conditions d'accès et les modalités d'attribution de l'aide d'urgence aux victimes de violences conjugales.

Dans sa première mouture, le texte ne prévoyait pas d'inclure cette disposition, qui est pourtant automatiquement proposée aux bénéficiaires du RSA aujourd'hui. Je me félicite donc de ce que la commission ait ajouté cette précision, qui figurait d'ailleurs dans le texte de ma proposition de loi relative à une aide financière d'urgence en direction des victimes de violences conjugales, déposée en 2021. Cette aide incombera au conseil départemental, lequel est déjà responsable de cette prise en charge pour les bénéficiaires du RSA, et consistera en une démarche d'accompagnement prenant en compte la situation globale de la personne et ses besoins : formation, santé, logement. Un tel dispositif proposé aux victimes de violences conjugales permettrait de limiter le risque d'un retour contraint au domicile conjugal, en favorisant l'accès à l'emploi et à une autonomie financière. Il me semblait important de souligner l'intérêt de cet ajout de la commission. La parole est

Mme Esther Benbassa. Cet amendement tend à s'inscrire dans la philosophie du présent texte. Quitter le foyer est l'une des décisions les plus difficiles. Le retour, quant à lui, est parfois inévitable. Cette proposition de loi encourage la victime à prendre l'initiative de la demande. Nous devons également nous assurer qu'elle lui permette d'être accompagnée jusqu'au bout de sa démarche. Il faut que le dernier lien soit rompu entre l'agresseur et l'agressé et que le parcours judiciaire de la victime soit complet. Le renoncement à la poursuite civile doit alors être un choix éclairé, délesté de l'emprise souvent persistante du conjoint violent. Cet amendement vise donc à préciser que le renoncement à la poursuite civile de l'agresseur doit être explicite. Quel

Le présent amendement tend à préciser le caractère explicite du renoncement de la victime. Cette précision n'apparaît pas comme utile et se trouve en réalité satisfaite. La caisse exercera les droits de la victime de manière subsidiaire. Il est donc clair, à ce titre, qu'elle informera expressément la victime de son intention d'agir en justice et que son action sera interrompue dès lors que la victime se constituera elle-même partie civile.

Madame la sénatrice Benbassa, vous souhaitez par cet amendement renforcer le principe de choix éclairé de la victime, pour aller jusqu'au bout de la démarche

Cet amendement de la commission tend à proposer une coordination avec le projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur (Lopmi), qui a été adopté par le Sénat. Il est ainsi prévu de créer la fonction d'assistant d'enquête pour seconder les officiers et agents de police judiciaire sur certaines tâches de procédure.

à votre disposition initiale, pour que nous avancions au mieux et dans le même état d'esprit : mieux protéger les victimes et leur permettre de reprendre leur autonomie. S'agissant de cet amendement, il semble semble nécessaire que les assistants d'enquête disposent d'une compétence d'attribution limitée, définie dans un nouvel article 21-3 inséré au code de procédure pénale, et sans autonomie d'intervention. Ce n'est qu'à cette condition essentielle que le Conseil d'État a admis a admis la validité de la disposition dans son avis du 10 mars dernier. En outre, il est prématuré d'ajouter des compétences aux assistants d'enquête alors que l'Assemblée nationale n'a pas encore examiné Le Sénat a d'ailleurs souhaité évaluer ce nouveau dispositif. Pour ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet

Si le dispositif fait preuve d'efficacité, il apparaîtra nécessaire de l'élargir aux caisses de la MSA, par équité de traitement entre les allocataires et par simplification de l'accès à l'aide pour les personnes victimes relevant du régime agricole, même si,

Le Houerou, pour explication de vote. Cette proposition de loi vise à mettre en place une avance universelle d'urgence à taux zéro, financée par la CAF, pour les victimes de violences conjugales.

le redis, un logement d'urgence situé au bord d'une quatre voies et sans accompagnement n'est pas une solution incitative à quitter l'enfer de la violence conjugale, une fois la crise aiguë passée. Or nous connaissons le phénomène du cycle infernal de la violence : la victime trouve des justifications aux violences